pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. Ma question s'adresse à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Il y a quelques semaines, à la suite du grand débat, le Président de la République a annoncé les grandes lignes d'un nouvel acte de la décentralisation. Une pièce au répertoire d'apparence classique pour nous, sénateurs, mais qui ne manque pas de susciter l'inquiétude des principaux acteurs : les collectivités locales. Aujourd'hui, cette pièce n'est pas encore à l'affiche, mais déjà les rumeurs bruissent et le ballet des suppositions donne quelque peu le tournis. Il s'agirait ainsi, je cite le ministre chargé des collectivités territoriales, « de faire une décentralisation qui reparte du citoyen, et non des élus ou de l'État Cette formule mériterait sans doute quelques explications. Madame la ministre, comme vous le savez, les collectivités locales ont en quelques années dû et su s'adapter au gré des réformes changements de périmètres des intercommunalités ou des communes, changements de compétences, délégations de compétences, baisses de dotations ont été réalisés dans des délais parfois très courts ou peu adaptés aux réalités locales.

ces incertitudes constituent des freins pour les projets locaux et pour l'investissement. Nous plaidons, à ce titre, pour un calendrier très précis. Nous plaidons pour que la question des moyens et de la fiscalité locale soit examinée en même temps. Nous plaidons pour que les collectivités soient confortées et mieux identifiées dans leurs rôles. Nous plaidons pour la préservation d'un maillage de proximité. Quel calendrier envisagez-vous ? Quelle méthode proposez-vous ? Quelle France des territoires voulez-vous ? La parole

clairs : responsabilité, lisibilité et financement. C'est à mon sens le triptyque nécessaire. Sur ce fondement, j'entends identifier au sein de ces champs les compétences susceptibles d'être confiées aux collectivités territoriales. Cette évolution se fera, bien entendu,

commun et de débattre avec les élus locaux. Au-delà de ces éléments de méthode, ce nouvel acte de décentralisation devra permettre de définir également la politique de contractualisation avec les collectivités locales dans les matières qui le nécessitent. J'ajoute que que nous discuterons du droit à la différenciation dans la réforme constitutionnelle à venir. Ces chantiers doivent s'articuler avec l'existant,

Le 9 mai dernier, le Conseil constitutionnel a rendu une décision historique en validant de manière incontestable la première mise en oeuvre d'un référendum d'initiative partagée. Ainsi, la privatisation d'Aéroports de Paris, bradage d'un service public national, sera soumise au vote de nos concitoyennes et de nos concitoyens. en oeuvre de cette procédure revêt tellement d'embûches que, en 2008, lors de son inscription dans la Constitution, personne ne croyait vraiment à sa réalisation. Il aura fallu l'exaspération suscitée par la politique d'Emmanuel Macron, un ultralibéralisme désordonné et dogmatique, pour permettre de franchir la première étape. Maintenant, 4,7 millions d'électrices et d'électeurs doivent approuver cette procédure référendaire pour que le cheminement démocratique se poursuive. monsieur le ministre de l'intérieur, qui, selon l'article 3 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013, devez mettre en oeuvre, « sous le contrôle du Conseil constitutionnel, le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi » soumise à référendum. C'est pourquoi huit parlementaires, dont cinq présidents de groupe représentant deux cent vingt-six députés et sénateurs, ont souhaité vous rencontrer pour examiner avec vous les conditions de la plus large participation à cet événement citoyen. À ce jour et par courrier, vous avez refusé de les recevoir, les renvoyant au président du Conseil constitutionnel. Cette attitude est inacceptable, car c'est vous qui aurez la responsabilité technique et politique du bon déroulement de cette consultation ! Monsieur le ministre, est-ce l'excès de consultation du peuple qui mine nos institutions ou la remise en cause systématique des votes et des espérances populaires ?

Madame la sénatrice, rappeler ce bon principe de fonctionnement et rappeler que le ministère de l'intérieur n'a pas vocation à court-circuiter le Conseil constitutionnel dans la mise en oeuvre de la consultation citoyenne sur ce sujet, ce n'est nullement

qu'avant même que le Conseil constitutionnel prenne sa décision nous avions préparé les dispositions techniques pour pouvoir agir. Sa décision est aujourd'hui confirmée, et nous serons prêts, dans le délai d'un mois, pour ouvrir la consultation pendant les neuf mois qui seront nécessaires. La parole

pour le groupe socialiste et républicain. Dans dix jours, les Français éliront leurs députés européens. Le Gouvernement est massivement entré en campagne. Cela se voit : les ministres sont sur tous les fronts, dans tous les territoires. Cela s'entend : les belles paroles et les promesses se multiplient. On a ainsi entendu parler d'un « tournant vert » de M. Macron lors de la présentation de votre programme. Un tournant, car ce n'était pas, jusqu'à présent, votre plus grand marqueur politique, ni européen ni national. À l'échelle européenne, le vide de la dernière déclaration de Sibiu est l'exemple même du manque d'ambition concrète de la France sur le climat, alors que l'accord de Paris a été notre honneur en 2015. Si La République En Marche promet aujourd'hui une banque européenne du climat, le Président de la République, qui siège au Conseil européen, ne l'a jamais évoquée avec ses pairs en deux ans. Au niveau national, les trous dans la raquette sont également nombreux. Ne prenons qu'un exemple récent : la suppression annoncée d'un train pour transporter les fruits et légumes de Perpignan à Rungis. Résultat : 25 000 camions de plus par an sur les routes. sur les routes. On est loin du ! Votre programme évoque aussi un tournant social et démocratique. Des notions qui font écho au discours de la Sorbonne. C'était il y a un an et demi, et les actes se font toujours attendre. Pis, ce sont des signaux contraires qui ont été envoyés par le Président de la République lorsqu'il s'opposait en première ligne aux avancées sociales et démocratiques européennes, à l'image de la directive Lanceurs d'alerte malmenée et de la directive Congé parental torpillée par la France. Comment expliquez-vous, monsieur le ministre d'État, le décalage entre ce programme et ce que vous avez réalisé depuis deux ans ?

pour la réplique. L'Europe mérite mieux qu'un troisième tour de l'élection présidentielle. Vous vous présentez comme un rempart contre l'extrême droite. En fait, vous avez organisé un rencart avec Mme Le Pen Vous kidnappez le débat européen ! L'Europe doit tourner la page du libéralisme et changer de cap pour devenir véritablement écologique et sociale, avec une nouvelle majorité de gauche au Parlement européen.

Compte tenu de l'augmentation significative des agressions et de la difficulté à gérer cette violence, une réflexion s'est engagée pour tenter de trouver des solutions nouvelles, d'où le concept « d'unité pour détenus violents », dont la vocation est de resociabiliser des individus pour lesquels la prise en charge classique n'est plus adaptée.

L'établissement nordiste dispose d'une expérience forte en matière de prise en charge psychologique et, donc, d'un vrai savoir-faire, ce qui a permis d'accélérer le dispositif. Cette unité, que j'ai eu l'occasion de visiter la semaine dernière, permet d'accueillir une dizaine de ces « détenus violents » dans des cellules individuelles, pour un suivi très personnalisé par des psychologues, des conseillers pénitentiaires et des surveillants. n'entre pas dans le détail, mais le séjour ne doit pas dépasser neuf mois. En discutant longuement avec les acteurs du projet, j'ai ressenti une véritable motivation, une conviction forte sur l'opportunité de ce concept, qu'il convient d'encourager. Certes, il faudra du recul pour apprécier l'efficacité de ce dispositif récent. Quelles seront donc vos orientations, madame la garde des sceaux ? On évoque le développement d'initiatives identiques à Strasbourg ou Marseille.

nouvelle structure. Nous avons en effet décidé d'ouvrir à Lille-Sequedin cette année une unité pour détenus violents. Ce projet s'inscrit dans un cadre plus général, que j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer devant vous : construire dans nos prisons

2019 et il est assuré grâce à la loi de programmation pour la justice, que vous avez bien voulu adopter, mesdames, messieurs les sénateurs. En conclusion, je souligne que les personnels pénitentiaires, qu'il s'agisse des surveillants ou des psychologues, sont spécialement formés pour

ces héros du commando Hubert, qui, avec leurs camarades, ont sauvé des otages, touristes inconscients du danger qu'ils couraient dans cette région du Nord-Bénin. Ces soldats ont accompli un exploit. Ils l'ont payé de leur vie, mais ils ont montré ainsi que la France n'abandonne jamais ses enfants. Nous ne les oublierons pas, et nous pensons à cet instant à leurs familles, à leurs camarades de combat et à ces milliers de soldats qui, pour notre compte, combattent au Sahel pour assurer la sécurité de l'Europe tout entière. Laissons de côté les polémiques sur les conditions d'accueil de ces touristes à l'aéroport de Villacoublay ou sur la couleur de la carte du Quai d'Orsay. Chacun a son idée sur ces sujets, et notre hémicycle n'est pas le lieu des polémiques.

puisque des touristes irresponsables continueront sûrement à chercher l'aventure dans ces contrées dangereuses, n'est-il pas temps d'exiger de ces pays à risque une politique plus sévère d'octroi des visas touristiques pour ces zones infestées par le terrorisme ? ? Plus largement, pouvez-vous nous assurer que tout va être fait pour que nos soldats, qui payent déjà un très lourd tribut à la lutte contre le djihadisme, n'aient pas en plus à payer de leur vie

vigilance accrue. Celles et ceux qui souhaitent se rendre à l'étranger doivent donc consulter systématiquement les conseils aux voyageurs, et je rends hommage au centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, qui veille à leur meilleure information possible, en lien naturellement avec les opérateurs de voyage. Nous devons

reconnu qu'ils auraient peut-être dû suivre plus scrupuleusement un certain nombre de recommandations -, mais aussi des opérateurs, notamment des plateformes en ligne, que je réunirai dans les prochains jours. S'agissant de la

Ma question prolonge celle de notre collègue Christian Cambon. Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello sont allés au bout de leur mission, jusqu'au sacrifice de leur vie. Ils ont permis la libération de quatre otages, dont deux de nos compatriotes. Notre groupe s'incline devant le courage et la détermination de ces deux militaires d'exception. Nos pensées vont à leurs proches, à leurs familles et à leurs frères d'armes. Cet événement tragique remet au coeur de l'actualité la situation politique de l'Afrique de l'Ouest. L'heure n'est pas à la polémique, comme cela vient d'être dit, mais plutôt aux questionnements sur les éléments liés à la sécurité dans cette bande sahélo-saharienne, dont la superficie, je le rappelle, est équivalente à celle de l'Europe. Je Je m'interroge tout d'abord sur la force conjointe du G5 Sahel. Cette dernière n'est actuellement pas en mesure d'assurer totalement sa mission, à savoir la sécurité dans la zone des trois frontières du Tchad, du Mali et du Niger. Le sera-t-elle d'ailleurs un jour, compte tenu des difficultés qu'elle rencontre ? Il est évident que les groupes armés terroristes ont des connexions entre eux et se jouent de la stratégie du G5 Sahel. Je m'interroge ensuite sur l'action de la France et son engagement dans cette région du monde. Nos forces armées font au quotidien un travail remarquable mais la France semble bien seule, même si elle est aidée efficacement par ses alliés historiques que sont nos amis Britanniques et Américains.

et le fanatisme ? La lutte contre le terrorisme est un enjeu international. Quand pourrons-nous enfin compter sur un véritable engagement européen au Sahel ?

pour apporter des réponses de long terme à cette zone sahélienne déstabilisée par de nombreux actes terroristes.

multidimensionnelle. Elle doit être sécuritaire, comme vous l'avez rappelé, avec la montée en puissance de la force conjointe G5 Sahel. Les Européens ont investi 100 millions d'euros pour équiper

Madame la secrétaire d'État, aujourd'hui même se tient le DuoDay, initiative qui permet à une personne en situation de handicap d'être accueillie par un professionnel au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une association. Lancé par un ESAT du Lot-et-Garonne et soutenu par votre action résolue, cet événement a pris désormais une ampleur nationale. Plus de 12 000 duos se sont ainsi constitués pour cette quatrième édition. Le temps de cette journée, employeurs et personnes handicapées vont se rencontrer, échanger et travailler ensemble, croiser leurs expériences et leur vécu. L'objectif est de développer les opportunités d'insertion professionnelle en surmontant les préjugés qui freinent l'emploi des personnes handicapées. La tâche est immense, comme nous le rappelle la citation d'Albert Einstein reprise sur la plateforme DuoDay : « Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé Si nous devons nous féliciter de la mobilisation grandissante autour de cet événement, ce changement de regard doit absolument s'accompagner de la mobilisation de tous faveur de politiques particulièrement volontaristes. En France, 2,7 millions de personnes sont en situation de handicap et en âge de travailler. Le taux de chômage des travailleurs handicapés est de 19 %, et trois quarts des demandeurs d'emploi handicapés ont un niveau de qualification inférieur au bac. Aussi, madame la secrétaire d'État, pourriez-vous nous détailler l'action du Gouvernement en matière d'incitation à l'emploi direct, de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de sécurisation des parcours professionnels pour les personnes en situation de handicap ?

et Social Européen. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur. Les scandales sanitaires récurrents placent la question du bien manger au coeur des enjeux de santé publique. Un pan du sujet n'est jamais évoqué : l'articulation entre ordre public et continuité alimentaire. Par le passé, notre modèle agricole reposait sur le foncier nourricier et sur un aménagement du territoire local multifonctionnel. La sécurité alimentaire était une préoccupation des élus. Aujourd'hui, production et consommation ne sont plus territorialisées, et même les zones rurales sont « alimentairement » vulnérables, perfusées par le ballet des camions de la grande distribution. À l'heure des cyberattaques, du dérèglement climatique et du terrorisme, production et approvisionnement alimentaires ne sont pas analysés comme des risques stratégiques. Des signaux nous alertent pourtant. La moindre annonce de blocage routier vide les magasins, avant même toute pénurie, allant jusqu'à provoquer des émeutes, comme il y a peu en outre-mer. En cas de force majeure, le déficit en capacité de subvenir localement à l'un de nos besoins primaires, celui de se nourrir, est flagrant. Les populations ne sont pas préparées. Assurer un niveau minimum de sécurité d'approvisionnement alimentaire est un devoir pour les autorités, qui devraient pouvoir garantir une chaîne résiliente allant du foncier agricole nourricier jusqu'au consommateur. Cela doit nous interroger sur la souveraineté et la sécurité nationales, articulées autour des biens communs, alors que les pouvoirs publics perdent peu à peu la main sur des infrastructures d'intérêt vital comme les aéroports, le foncier agricole ou la gestion de l'eau. Il est urgent de s'en préoccuper.

points d'approvisionnement soient visés. Là encore, nos forces de sécurité intérieure ont fait la démonstration de leur capacité à libérer ces points quand cela était nécessaire, sans pour autant provoquer de tensions extrêmement graves. La parole

mais nous avons en commun de ne jamais accepter que des informations médicales et nominatives soient transmises à des personnes qui ne concourent pas directement aux soins. Il s'agit en effet d'une violation grave du secret professionnel. Le fichier Sivic est une procédure exceptionnelle déclenchée en cas d'afflux exceptionnel de victimes. Il a été détourné de son objet à l'occasion du mouvement dit des « gilets jaunes ». Du seul fait de leur participation à ce mouvement, des personnes ont vu des informations médicales et nominatives être collectées et transmises. L'AP-HP, après des déclarations successives, a fini par admettre la réalité des faits. Les signataires ont interpellé le Parlement. Madame la ministre, allez-vous diligenter une enquête indépendante sur ces faits ? Allez-vous désavouer et faire cesser cette collecte d'informations, qui ne respecte pas les conditions posées par la CNIL à la mise en oeuvre de Sivic ? Très bien

à répondre à une arrivée exceptionnelle de blessés lors d'un événement particulier. Il est activé lorsqu'un événement est susceptible de générer beaucoup de blessés et désactivé quand l'événement en question prend fin. À titre d'exemple, le système Sivic a été activé récemment lors de l'explosion liée à une fuite de gaz dans le IX arrondissement de Paris ou des inondations dans l'Aude.

aux hôpitaux et aux ARS en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Néanmoins, la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, l'a rappelé et répété : « Jamais nous n'accepterons que l'on demande aux soignants de ficher des gilets jaunes qu'ils soignent. Jamais, d'ailleurs, ils n'accepteraient. » Il y a eu un malentendu. Pouvoir repérer les victimes de blessures en marge de manifestations pour adapter le système de santé ne veut pas dire ficher les « gilets jaunes ». Lors des manifestations où Sivic a été activé, toutes les personnes en lien avec les manifestations- forces de l'ordre, journalistes, passants et manifestants -ont pu potentiellement être entrées dans le fichier, sans distinction. Nous avons demandé à la direction compétente du ministère de la santé, à l'AP-HP et aux ARS de faire acte de transparence, notamment sur le fonctionnement de Sivic. Il faut conclure ! C'est ainsi qu'une inspection commune de l'ARS Île-de-France et de l'AP-HP est diligentée afin d'évaluer s'il y a eu des dysfonctionnements et pour s'assurer que ce fichier sera désormais strictement strictement constitué d'informations.

Les Républicains. Ma question s'adressait à Mme la ministre des solidarités et de la santé. Madame la ministre, vous le savez, l'une des préoccupations majeures des Français concerne l'accès aux soins, et plus spécifiquement la possibilité de trouver un médecin à proximité de leur lieu de vie. Il existe sur le territoire national des régions entières où cette difficulté d'accès pose un grave et réel problème de santé publique. La région Centre-Val de Loire et le département du Loiret sont parmi les plus défavorisés en nombre de médecins par habitant. Un rendez-vous chez un cardiologue, c'est un an ; pour consulter un ophtalmo. Il faut six mois pour rencontrer un allergologue ou un gynécologue, et, pour un nouvel arrivant dans l'Orléanais, il est quasiment impossible de trouver un généraliste. La région, le département et les communes se sont mobilisés depuis longtemps, avec constance et ténacité, pour proposer des solutions. En vain, car, si les structures existent, encore faut-il trouver les praticiens pour les remplir même constat peut être effectué dans de très nombreux autres départements. Outre mes collègues du Loiret, Rémy Pointereau, sénateur du Cher, s'associe à cette question qu'il souhaitait lui aussi poser.

Tant mieux pour les grands centres urbains tels que Paris, Lyon, Aix-en-Provence, Marseille et quelques autres, où le nombre d'admissibles progresse sensiblement. Mais qu'en est-il des facultés sièges de territoires plus ruraux tels que Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Poitiers, Reims et Tours, notamment ? Le ! Au Au total, on constate, pour cette dernière année d'existence du, une stagnation inquiétante pour dix-sept des trente facultés de médecine de la métropole. Ce qui nous scandalise, c'est l'absence de prise en compte du problème dramatique que constitue la désertification médicale dans la définition du nombre d'étudiants admis à suivre des études de médecine.

la lutte contre la désertification médicale est au coeur du plan Ma santé 2022 et du projet de loi Santé, dont l'examen vient de commencer au Sénat en commission.

Quelles propositions seront faites dans le cadre du projet de loi Santé ? Il s'agit de permettre à des jeunes de démarrer leurs études médicales dans tous les territoires, et non plus seulement dans les métropoles où se situent des CHU.

brûlot antisémite déroulant sa haine à longueur de pages. À la suite d'une intervention conjointe de collègues britanniques et de la Fondation des musulmans contre l'antisémitisme, nous avons pu obtenir sa suppression par Google le 11 mai dernier, mais l'application est toujours disponible

Or ce centre, proche des Frères musulmans, a été fermé par les autorités mauritaniennes, car il enseignait un islam radical. Lors d'une vidéoconférence, le cheikh Dedew, connu pour prêcher un islam radical, antisémite, a reproché aux musulmans d'avoir exprimé leur tristesse lors de l'incendie de Notre-Dame.

chef de file du G5 Sahel, que nous soutenons avec nos troupes dans cette région ? Pouvez-vous faire interdire cette manifestation et cette application ?

La Commission européenne paraît déterminée à conclure au plus vite un accord commercial avec le Mercosur, c'est-à-dire avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Le ministre brésilien du commerce, Lucas Ferraz, vient d'ailleurs de déclarer que la conclusion d'un accord « n'a jamais été aussi proche

La Commission fait des choix de plus en plus singuliers dans le monde. On peut légitimement se demander s'il est raisonnable d'envisager de brader notre souveraineté alimentaire. N'y a-t-il pas une contradiction à faire de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité et à envisager « en même temps l'importation de volumes de viande ne répondant à aucune demande, alors que la sagesse et la cohérence devraient nous conduire à choisir une autre voie ? Monsieur le ministre, allez-vous défendre les intérêts des éleveurs et des consommateurs ?

Le Président de la République s'est entretenu samedi dernier avec le président Juncker. J'ai moi-même travaillé de longues heures avec le commissaire Hogan. Notre position est claire

détriment de notre agriculture. La France est opposée à cet accord, parce qu'il se ferait au détriment de nos standards sanitaires. La France est opposée à cet accord, parce qu'il se ferait au détriment de nos standards alimentaires. Enfin, la France est opposée à cet accord, parce qu'il se

sa mairie, ce dernier service de proximité dans de très nombreuses communes, là où bat le coeur de notre démocratie. Désormais, cette démarche ne peut se faire que dans les mairies équipées d'une station d'enregistrement. Dans l'Oise, sur 679 communes, seules 27 en sont équipées, soit moins de 4 il ne faut surtout pas être pressé, car les délais d'attente peuvent dépasser les trois mois, non pas pour obtenir ses papiers, mais simplement pour déposer ses photos et compléter son dossier ! Ce passage à l'ère biométrique n'aura fait gagner ni temps, ni argent, ni énergie.

Bien des élus locaux regrettent de ne plus accueillir en mairie leur population à l'occasion du renouvellement de leurs titres d'identité. C'était parfois l'unique moment où ils pouvaient rencontrer leurs administrés, l'unique occasion pour certains habitants de se rendre en mairie.

réplique. Un ancien Président de la République avait promis un choc de simplification ; un autre avait demandé qu'on arrête d'emmerder les Français. Force est de constater qu'ils n'ont pas été entendus ! Pour conclure, je vous laisse méditer la devise d'une belle commune de l'Oise, Pierrefonds : « Qui veult peult

La séance est reprise.

ne seront pas prises en compte dans le calcul de l'objectif national d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales. Si je suis favorable sur le fond aux dispositions que tendent à prévoir ces amendements, elles relèvent d'une circulaire du ministre du budget, qui fixe le périmètre des dépenses concernées.

pour les communes et leurs groupements est estimé à 150 millions d'euros, selon les calculs de certains syndicats, la compensation de l'État, qui repose sur des évaluations encore imprécises, serait d'environ 50 millions d'euros en direction des maternelles privées, un peu plus s'agissant du remboursement des forfaits des maternelles publiques.

du rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale. En outre, en application de l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative sur l'évaluation des charges établit à l'intention du Parlement un bilan annuel de l'évolution des charges transférées aux collectivités locales.

à M. le ministre. L'article 4 dispose que l'instruction obligatoire peut être dispensée à titre dérogatoire dans les jardins d'enfants. Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait une dérogation de deux ans. Votre Votre commission a souhaité rendre cette dérogation pérenne. Une telle proposition présente, selon le Gouvernement, un risque de rupture d'égalité, notamment vis-à-vis des écoles privées hors contrat.

et de préparer les éventuelles évolutions et reconversions professionnelles de leurs employés. Plusieurs voies d'évolution articulées au développement des modes d'accueil du jeune enfant sont possibles pour les jardins d'enfants. est de demeurer un jardin d'enfants, en se recentrant sur la tranche d'âge de 2 à 3 ans et être ainsi une passerelle douce vers l'école- cela peut être très fructueux.

en école maternelle hors contrat avec un projet éducatif et pédagogique défini, puis, le cas échéant, et selon les dispositions en vigueur, en école maternelle sous contrat. Les évolutions de ces structures doivent être analysées au cas par cas, en fonction des projets propres portés par les jardins d'enfants existants- par exemple, ceux qui ont des méthodes éducatives alternatives, ceux qui pratiquent le bilinguisme, etc. -, mais également en fonction des besoins locaux en matière d'accueil préscolaire et scolaire. Chaque structure pourra ainsi évoluer vers la forme juridique qui lui correspond le plus. L'État, au travers des plans de formation dédiés pour les personnels, pourra accompagner certaines structures qui le souhaiteraient vers leur transformation en école maternelle publique. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement propose, avec cet amendement, de rétablir une dérogation limitée dans le temps pour les jardins d'enfants. Nous optons pour un délai plus important que celui qui avait été adopté par l'Assemblée nationale, en passant de deux à trois ans. Durant cette période de trois années, ces établissements feront l'objet d'un contrôle de la part des services académiques, afin de vérifier que l'instruction, telle qu'elle est prescrite nationalement, y est effective. Les jardins d'enfants sont aujourd'hui un type particulier d'établissement d'accueil du jeune enfant. C'est évidemment important de respecter ce qu'ils ont accompli. Je suis le premier à reconnaître qu'il y a des choses très positives dans le bilan que l'on peut en faire. Comme dans d'autres Comme dans d'autres situations, il faut, je crois, avoir la démarche de garder ce qui est positif, de faire évoluer ce qui l'est moins, de sorte que les jardins d'enfants profitent de ce nouveau contexte pour apporter leur expérience et se transformer selon l'une des modalités que j'ai indiquées.

sans aucune réflexion, sans aucune audition. On se demande même si le ministre n'a pas découvert les jardins d'enfants, qui sont dans le code de la santé publique, au hasard de ce projet de loi. Monsieur le ministre, ce système fonctionne et a fait ses preuves.

a effectivement une tradition de jardins d'enfants extrêmement importante. Ils fonctionnent bien. Votre objectif, monsieur le ministre, c'est que les enfants, dès l'âge de 3 ans, soient pris en charge dans une structure dans le but d'y recevoir une instruction. Or il s'avère que ces jardins d'enfants, comme l'a dit David Assouline, ont apporté cette instruction sans que personne les critique.

de votre prise de position. Monsieur le ministre, au lieu d'une mise à mort en deux ans, vous proposez une mise à mort en trois ans. Franchement, c'est déplorable ! Madame Cartron, ne soyez pas méprisante ... Mais non ! ... à l'égard d'un travail qui est fait depuis un siècle.

que la commission de la culture ait adopté mon amendement, car elle a compris quel est le rôle essentiel de ces jardins d'enfants dans un certain nombre de territoires. Vous avez quand même là 10 000 jeunes

a été rejetée, malgré un vote qui frôlait l'unanimité. Vous en connaissez les conséquences, monsieur le ministre, et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, le Sénat vous appelle encore à la sagesse. Ce Sénat des territoires ; ce Sénat qui est composé d'anciens élus locaux, voire d'élus locaux toujours en exercice- c'est mon cas - ; ce Sénat composé de personnes qui ont été maires, voire ministres et qui ont cette connaissance de la réalité des territoires. Pour ma part, j'habite une région où chaque parcelle d'activité vaut de l'or.

ans. En Bretagne, nous n'avons pas de jardins d'enfants, parce que c'est l'école privée catholique qui a proposé de scolariser tous les enfants, parfois même à l'âge de 2 ans. J'entends parler de décentralisation, de différenciation. Je suis donc gênée que l'on ne prenne pas en compte des expériences très positives qui ont été conduites dans des territoires et qui correspondent à une culture, à une histoire

les jardins d'enfants sont payants, les écoles privées hors contrat ou sous contrat aussi. Certains ont l'air de découvrir quelque chose de nouveau, mais il y a longtemps que notre système fonctionne ainsi. Enfin, nous avons voté hier à l'unanimité l'abaissement

Je ne suis pas en très grand désaccord avec une bonne partie de ce qui a été dit par les uns et par les autres. Si vous m'avez écouté, reconnaissez que je n'ai cessé de dire que nous devions suivre la voie la plus pragmatique. Je ne veux absolument pas la mort des jardins d'enfants et encore moins mettre au chômage ceux qui y travaillent.

Il y a des choses excellentes qui s'y passent, et je les salue sans aucun problème. Ils peuvent même être, à certains égards, un modèle pour l'école maternelle. Et puis, il y a des choses qui ne vont pas. C'est très hétérogène d'un endroit à l'autre. C'est vrai ! Il me semble même, monsieur Assouline, que le maire de Paris avec qui vous avez travaillé, Bertrand Delanoë, avait envisagé

mon but n'est certainement pas de « supprimer » les jardins d'enfants. Ce mot est beaucoup trop fort. Nous voulons une période de transition pour que les jardins d'enfants puissent maintenir ce qui va bien et s'améliorer sur ce qui ne va pas.

On aura ainsi un continuum jardin d'enfants-école maternelle qui peut être excellent. Je citais hier le cas d'Arras, où il y a une très bonne coopération entre les personnels municipaux de la petite enfance et les personnels de l'éducation nationale. C'est très souhaitable d'arriver à ce type d'organisation. Je n'ai aucun problème à m'associer à l'hommage que vous avez rendu, monsieur le rapporteur,

a toutes les chances d'exister encore demain. Simplement, il aura vécu des transformations qui l'auront tiré vers le haut, et je suis tout à fait prêt à donner des garanties en la matière. Je termine mon intervention

Ces structures sont soumises à l'autorisation des représentants de l'État à l'échelon local. Il ne devrait donc plus y avoir de création de nouvelles structures sous cette forme juridique, mais nous devons nous en assurer. Tel est l'objet de cet amendement du Gouvernement. Comme vous le comprenez, il s'agit aussi d'éviter- c'est l'une des raisons

dont le statut se rapproche de celui des jardins d'enfants, de bénéficier d'une dérogation de deux ans pour dispenser l'instruction obligatoire aux enfants de trois à six ans qui y sont inscrits, et ainsi leur permettre de se mettre en conformité avec le droit dans ces deux ans afin de continuer à dispenser l'enseignement obligatoire au-delà de cette période transitoire. Certaines structures recevant des enfants entre deux mois et six ans seraient exclues du dispositif de dérogation accordé aux jardins d'enfants, adopté à l'article 4 par la commission de la culture du Sénat. Or nombre de ces établissements, présents en Alsace notamment et en Meurthe-et-Moselle, le département de Véronique Guillotin, proposent un circuit éducatif fondé sur le bilinguisme. Les enfants accueillis doivent pouvoir continuer à accéder à une telle formation,

Me voilà maintenant accusé de vouloir être une sorte d'extrémiste de l'école maternelle ! C'est vrai ! Sans doute est-ce le lot d'un gouvernement qui se situe là, au centre d'un hémicycle, de se prendre ainsi du vent à droite, du vent à gauche et, à la fin, du vent des deux côtés, dans une sorte de

Le scrutin est ouvert.

République. Le nombre d'enfants instruits en famille est en très nette progression. En dix ans, entre 2007 et 2017, la hausse a été spectaculaire, puisqu'elle a été de 122 %. Aujourd'hui, plus de 30 000 enfants sont instruits en famille. Cette progression me paraît quelque peu préoccupante, d'autant que la proportion d'enfants inscrits au CNED en classe à inscription réglementée décroît fortement, pouvant faire craindre des situations de radicalisation. À cet égard, j'ai été interpellée par les propos de l'avocat de l'école privée hors contrat d'Échirolles, que vous entendez fermer, monsieur le ministre, car « d'inspiration salafiste ». Il dit : « Les parents de ce quartier prioritaire ne voulaient pas ou plus mettre leurs enfants à l'école publique. Sur la centaine d'élèves inscrits à cette école, une trentaine était auparavant scolarisée à domicile. » On le voit, nous sommes confrontés à un sujet préoccupant, qui prend de l'ampleur. Aussi, je me réjouis que le présent projet de loi s'en saisisse de nouveau. J'approuve le principe de mise en demeure de scolariser l'enfant en cas de refus réitéré de se soumettre au contrôle obligatoire. En effet, aujourd'hui, les services de l'État sont dépourvus de solution immédiate. Quant aux lieux du contrôle, certains parents s'appuient sur l'ambiguïté de la loi pour opposer un refus aux inspecteurs de l'éducation nationale. S'il est nécessaire de préciser que ce sont bien les services de l'État qui déterminent les modalités du contrôle, il est important de réaffirmer le principe du contrôle sur le lieu de l'instruction, à l'inspecteur d'apprécier l'environnement, ainsi que les méthodes et les ressources utilisées et donc de mieux appréhender les dérives potentielles. Comme je l'avais déjà indiqué lors du débat sur la loi Égalité et citoyenneté, outre les aspects juridiques, se pose la question fondamentale des contrôles. Il est encore aujourd'hui regrettable qu'une part significative des enfants instruits à domicile ne fasse l'objet d'aucun contrôle. Environ un quart des élèves n'a pas fait l'objet d'un premier contrôle. Il y a plus grave, monsieur le ministre, mais les derniers chiffres dont je dispose sont ceux de 2014-2015. À ces dates, À ces dates, 40 % des premiers contrôles d'instruction en famille considérés comme insatisfaisants n'avaient donné lieu à aucun second contrôle, alors que la loi l'impose. L'État doit allouer des moyens nécessaires à l'exécution de la loi, pour éviter toute dérive. Je connais votre engagement et votre détermination. Disposez-vous de chiffres plus récents nous permettant de mesurer les évolutions des contrôles de l'instruction en famille

Cette expansion a malheureusement mis en lumière les failles de l'identification et du contrôle de l'instruction à domicile, qui peuvent également être détournés par des mouvements prônant des valeurs contraires à celles de la République. Or un certain nombre d'élèves échappent encore au suivi de l'État ou des services sociaux. Retirés de l'école, sans être déclarés comme étant instruits à domicile, absents des registres ou mal instruits, ces enfants peuvent parfois être dans des situations à risque. Aujourd'hui, l'identification, le contrôle, le suivi et la connaissance des enfants identifiés comme étant instruits à domicile sont clairement insuffisants. C'est pourquoi, en s'inspirant d'une proposition de la mission flash de l'Assemblée nationale du 18 juillet 2018 concernant la déscolarisation, ma collègue Nathalie Delattre a déposé un amendement visant à améliorer le suivi et l'identification au niveau national des enfants non scolarisés en leur attribuant à tous un numéro d'identification national élève, l'INE, dès l'âge de la scolarité obligatoire, soit 3 ans. Jugé irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution, cet amendement aurait pourtant permis d'élargir l'attribution d'un numéro d'identification national élève à tous les enfants, en incluant ceux qui sont scolarisés à domicile. Il convient de mettre en place un traitement des données à caractère personnel couvrant l'ensemble de la population en âge scolaire pour contrôler le respect de cette obligation d'instruction. Pour cela, monsieur le ministre, vous avez déclaré devant le Parlement qu'« il suffisait de modifier la portée d'outils informatiques déjà existants par voie réglementaire ». C'est la raison pour vous demander si, avec le Gouvernement, vous entendez bien agir sur cette mise en place. La solution est simple, il suffit juste d'en avoir la volonté et si possible rapidement. La parole

Françoise Gatel, en précisant que j'ai été rapporteur d'une commission d'enquête au Sénat sur l'évolution de la menace terroriste en France et en Europe. Dans ce cadre, nous avons auditionné de nombreuses personnalités, parmi lesquelles certains de vos collègues ministres et des représentants de l'éducation nationale. Sur la question du contrôle des nombreux enfants déscolarisés dans certains quartiers, le problème était non pas le contrôle en lui-même, mais les capacités des contrôleurs à se rendre sur place. On nous a répondu textuellement qu'ils ne contrôlent pas et ne se rendent pas dans les familles non pas parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, mais parce qu'ils ont peur. Je voulais profiter de cet instant

Comme on le dit très souvent, l'éducation permet d'éviter certains écueils. Comme vous, je tiens à ce que l'éducation nationale, au-delà de sa fonction d'ascenseur social, protège nos enfants de certaines dérives. Ces contrôles sont très importants. Or, bien souvent, les familles ne sont pas contrôlées.

Actuellement, le maire a la responsabilité de mener le contrôle visant à vérifier les conditions de vie des enfants et à établir les raisons ayant motivé ce choix d'instruction. Le contrôle de la mairie doit aussi déterminer s'il est bien donné aux enfants une instruction compatible avec leur état de santé. un certain nombre de maires, par manque d'information ou de moyens, ne conduisent pas ces contrôles, parfois délicats à mener, notamment en raison du sentiment d'intrusion qu'ils peuvent générer dans les familles. de la circulaire n° 2017-056 du 14 avril 2017 relative au contrôle de l'obligation scolaire et du guide interministériel du 27 novembre 2017 sur le rôle des acteurs locaux dans le cadre de l'instruction dans la famille, l'obligation pour les maires d'assurer ce contrôle reste mal connue des élus locaux et soulève l'incompréhension des administrés.

les résultats du contrôle pédagogique.

Laborde s'agissant de notre capacité numérique, ce qu'on appelle le DNE, cet identifiant numérique, sera prêt

voire à un harcèlement. Il est indispensable que le contrôle tienne compte de cette anxiété ou du retard accumulé en établissement avant le début de l'instruction dans la famille.

déterminées unilatéralement par l'inspecteur le jour du contrôle, selon la première phrase de l'alinéa 5, mais aussi déterminées par décret, selon la troisième phrase. Pour éviter des contrôles hétérogènes en fonction des inspecteurs, et donc des litiges dus au non-respect par l'inspecteur du décret d'application, il est souhaitable que les modalités de contrôle soient uniquement définies par décret. Quel est l'avis de

il s'effectue, en affirmant clairement qu'il revient à l'État de déterminer le lieu, la date et le contenu du contrôle de l'enseignement, ce qui me semble de bonne administration.

à vos déclarations relatives à la loi Gatel, monsieur le ministre, j'entends bien que vous considérez qu'il vous manque un certain nombre d'instruments légaux qui vous permettraient d'intervenir.

L'amendement n° 130 vise, quant à lui, à fixer un délai de deux mois après la communication des résultats du second contrôle pour mettre en demeure la famille de scolariser son enfant. Un tel délai ne m'apparaît pas pertinent, car il me semble beaucoup trop long. Si le second contrôle est insuffisant, la mise en demeure doit, selon

: La parole est à M. Philippe Mouiller. Je présente cet amendement au nom du président de notre groupe, M. Bruno Retailleau. Un amendement adopté en commission au Sénat a exclu les établissements privés hors contrat du champ des établissements dans lesquels la famille peut scolariser son enfant dans le cadre d'une mise en demeure de l'inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire. scolaire. Or nous considérons qu'une telle distinction n'est pas justifiée et est de nature à créer une rupture d'égalité, dès lors que l'établissement d'enseignement privé hors contrat est légalement ouvert et qu'il est contrôlé par l'État. Cela reviendrait également à considérer que, par principe, les établissements d'enseignement hors contrat ne dispensent pas un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire telle qu'elle est définie à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation. De ce fait, cette disposition porte atteinte au droit de choisir l'instruction de son enfant, qui est une composante de la liberté de l'enseignement. Le présent amendement vise donc à la supprimer. Quel est

assez mal à l'aise dans l'exercice de leurs fonctions. Je sais, monsieur le ministre, que vous avez mis en place, à l'exemple de ce qui s'est fait dans l'académie de Versailles, un accompagnement et une formation à destination de ces inspecteurs. Ces contrôles doivent être faits de manière neutre

peuvent être sanctionnés : on peut les contraindre à scolariser leurs enfants dans une école publique. Ce n'est pas une infraction à la liberté d'enseignement : c'est obliger quelqu'un à réparer une faute qu'il a commise. La parole est à Mme Josiane Costes, pour explication de vote.

contrat est imparfait : il nous faut véritablement privilégier l'intérêt de l'enfant et faire en sorte qu'il soit scolarisé dans des établissements publics ou privés sous contrat.

contre cet amendement.

qui est inadmissible, qui pose problème, qui met en danger des enfants, je peux vous assurer qu'il est très difficile de la traiter. Je suis moi-même maire d'une commune qui a été face à une telle situation : une école hors contrat

la commission ? À la différence de l'absentéisme, la méconnaissance d'une mise en demeure d'inscrire son enfant dans un établissement scolaire est pénalement réprimée. La peine encourue est de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Elle peut être assortie de peines complémentaires, comme l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ou l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.

Il ne s'agit pas de chiffres ; il s'agit d'enfants et de leur rapport à la scolarisation ou, plutôt, à l'instruction. Ce qui a motivé la commission est la chose suivante : il peut y avoir un blocage entre l'inspecteur et la famille. Le fait d'avoir un second regard est une pratique qui est très fréquente à l'éducation nationale ; je peux en témoigner. En général, quand il y a blocage,

monsieur le rapporteur, et exige un projet pédagogique. Le Sénat s'était prononcé clairement contre cela afin d'éviter un contrôle d'ordre purement pédagogique, ce qui serait contraire à la liberté de l'enseignement. Nous ne sommes pas naïfs pour autant. C'est pourquoi à adopter des amendements présentés par Françoise Gatel et par le Gouvernement qui apportent des retouches au dispositif de la loi Gatel afin de le rendre plus opérationnel.

que tout porteur d'un projet d'établissement scolaire doit demander une autorisation de recevoir du public avant de déposer sa déclaration d'ouverture d'un établissement scolaire.

s'il répond à l'obligation d'instruction, à l'obligation de formation ou aux deux. C'est la raison pour laquelle l'établissement sera tenu de déclarer qu'il entend préparer ses élèves à des diplômes ou emplois différents de ceux dont il avait, le cas échéant, déjà fait part à l'administration.

persistantes à l'ordre public dans un établissement hors contrat, à créer un délit et une injonction de rescolarisation et à faciliter le contrôle du régime des incapacités pénales pour exercer dans ces établissements. Comme Comme nous l'avons évoqué lors de l'examen des amendements précédents, la loi du 13 avril 2018 a trouvé un point d'équilibre entre la liberté de l'enseignement et les garanties que l'État doit aux enfants pour qu'ils bénéficient de manière effective du droit à l'éducation. Cet équilibre est efficace, il doit être conservé ; l'amendement que je vous présente le maintient. Sur le plan formel, il est apparu que la mention des seuls titres des professeurs, dont la liste est transmise chaque année au recteur, n'était pas toujours bien comprise par les déclarants au sein des établissements. Cette mention n'a pas constitué un obstacle à la mise en oeuvre de la loi, mais il est apparu plus simple et plus clair d'ajouter à la mention des titres celles de l'identité, de l'âge et de la nationalité. nationalité. Sur le fond, cet amendement conforte et prolonge la garantie déjà offerte aux enfants quant au respect de l'ordre public dans les établissements hors contrat. Le premier alinéa de l'article L. 442-2 prévoit déjà

au moyen de l'injonction de rescolarisation, dans la même logique que celle déjà en vigueur lorsqu'il y a persistance à ne pas respecter le droit à l'éducation des enfants. Pour ces raisons, je vous invite à voter cet amendement, qui ne crée pas un nouveau contrôle ni ne remet en cause la liberté pédagogique. Il permet simplement de tirer toutes les conséquences des contrôles existants.

conséquences. S'agissant de ces nouveaux établissements, trois d'entre eux se trouvaient en situation d'illégalité, notamment pour des atteintes portées à l'ordre public ou du point de vue de la protection de l'enfance et de la jeunesse. Ces trois établissements ont fait l'objet d'une procédure en vue de leur fermeture.

afin de recenser les enfants scolarisés dans sa commune et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire. Actuellement, l'article L. 131-6 du code de peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales, ainsi que par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement. d'allocations familiales, notre commission a décidé d'ajouter des données transmises par les services fiscaux. Autant la politique éducative est liée à celle des prestations familiales, autant on ne voit pas bien en quoi la transmission par les services fiscaux des déclarations d'impôt des familles participerait de la scolarité obligatoire et en quoi ces données présenteraient un quelconque rapport ou intérêt avec l'obligation d'instruction. Bien au contraire, il me semble néfaste que les maires aient communication de la situation fiscale de leurs administrés qui ont des enfants en âge scolaire. Il y va

La mission flash de nos collègues députées Anne Brugnera et George Pau-Langevin a mis en évidence les difficultés des maires, particulièrement en ville, à recenser effectivement les enfants en âge d'être

La loi investit le maire d'une mission de mise en oeuvre et de contrôle de l'obligation scolaire des enfants de sa commune. L'article 5 lui permet, s'il est témoin d'un manquement aux obligations des familles en matière d'obligation scolaire, de saisir le procureur de la République. Ces dispositions ne visent pas le contenu de l'enseignement dispensé dans le cadre de l'instruction à domicile, mais d'autres délits prévus par le même chapitre : le fait, pour la famille, de ne pas procéder à la déclaration d'instruction dans la famille ; le fait de ne pas se conformer aux obligations d'assiduité scolaire ; le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure de scolariser son enfant prévue par le code de l'éducation. Il me paraît parfaitement légitime que le maire puisse, de sa propre initiative, saisir le procureur de la République en la matière. Il s'agit de la reconnaissance légitime de ses prérogatives. C'est pourquoi je vous invite, ma chère collègue, à retirer cet amendement.

Darcos. Aux termes de l'article 5 , les maires sont désormais encouragés à effectuer un signalement s'ils suspectent une insuffisance d'instruction, c'est-à-dire à détecter les enfants non scolarisés et non déclarés en instruction en famille. Or cette rédaction n'est pas claire. C'est pourquoi cet amendement vise à préciser que le maire a uniquement pour mission de référencer, et non celle de juger de l'effectivité de l'instruction.

doivent se faire au sein des établissements d'enseignement public par le personnel enseignant de ces établissements. Actuellement, les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille sont évalués lors du contrôle pédagogique avec des exercices écrits et oraux adaptés à leur âge. Rien n'est prévu quant aux modalités de mise en oeuvre de ces exercices et quant au personnel chargé de les évaluer. Organiser ces contrôles au sein des établissements d'enseignement public

des conditions d'ouverture des établissements privés et de procéder aisément à un retrait de l'autorisation en cas d'infraction. L'autorité académique sera chargée d'instruire le dossier procureur de la République ... -des suites données à la demande d'autorisation. Le régime déclaratif n'est pas entièrement satisfaisant. La création d'un régime d'autorisation permettrait de suspendre ou de retirer l'autorisation. Je tiens à rappeler que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur l'incompatibilité d'un tel régime avec la liberté d'enseignement. Cette liberté, principe à valeur constitutionnelle, emporte certes des droits, comme celui d'établir un projet pédagogique alternatif ou de percevoir un financement public dans certaines conditions pour les établissements sous contrat, mais elle a toujours comporté des limites qu'il est loisible au législateur de fixer.

La France est en retard quant à leur prise en charge. La majorité d'entre eux est au collège ou au lycée. Leur situation génère beaucoup de stress et crée énormément de difficultés chaque jour. Pis, certains se déscolarisent petit à petit. Ce n'est donc pas un élément à prendre à la légère. Les pouvoirs publics doivent leur venir en aide, il y a urgence ! C'est pourquoi j'avais proposé des pistes pour faciliter leur quotidien. Certaines de ces mesures sont d'ailleurs déjà en place pour des jeunes qui sont dans d'autres situations, par exemple les enfants et adolescents handicapés. Ainsi, mon amendement entendait répondre à plusieurs objectifs. J'en citerai quelques-uns : permettre l'inscription dans une école ou un établissement au plus proche de leur domicile, ce qui ne coûte rien assurer un parcours de formation adapté, en créant un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires et en évaluant leurs compétences et leurs besoins ; permettre permettre des aménagements aux conditions de passation des examens ou des concours de l'enseignement scolaire et supérieur avec un temps supplémentaire accordé ; former les enseignants et les personnels à l'accueil et l'éducation des jeunes aidants, formation qui comporte notamment une information sur la lutte contre la stigmatisation

L'esprit de ce projet de loi est de donner une meilleure justice sociale à tous et de permettre l'égalité des chances pour tous les enfants, y compris ceux qui sont en situation de handicap. Le statut des accompagnants est valorisé

Les accompagnants ne sont plus recrutés sous contrat unique d'insertion, ce qui met fin au recrutement des contrats aidés. Les établissements font aussi l'objet de réformes dans le cadre du présent article. Ils sont le lieu central pour l'instruction de nos enfants. Il convient de mieux les penser afin que nous soyons véritablement fiers d'avoir une école inclusive.

C'est pourquoi le dispositif des pôles inclusifs d'accompagnement localisé, expérimenté depuis la rentrée de 2018, aura une accroche législative dans ce projet de loi. Ces pôles coordonneront les moyens humains dédiés à l'accompagnement des élèves en situation de handicap au sein des écoles. Ils permettront ainsi de mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers ; nous sommes convaincus que l'aide mutualisée peut contribuer, au même titre que l'aide individualisée, à la réussite des élèves. Avant de terminer mon propos, je souhaite apporter un témoignage, qui renforcera notre argumentation.

Nous reprendrons certainement à notre compte toutes les propositions qui seront faites ; le texte va dans le bon sens, il faut simplement continuer nos efforts.

ce sujet. Il y a évidemment beaucoup à faire, et, on le voit, rentrée après rentrée, les choses sont de plus en plus chaotiques du point de vue de l'accueil, notamment depuis la suppression d'un grand nombre d'emplois aidés. Il y a donc besoin de créer un statut véritablement attractif pour répondre à la crise du recrutement

des notifications ou ne pas reconduire des accompagnements, en attendant les modifications législatives ; c'est évidemment scandaleux. Il est même parfois précisé qu'il faut éviter de mettre les familles au courant,

M. Olivier Paccaud, sur l'article. Avec la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la scolarisation des élèves handicapés dans le milieu scolaire est devenue un principe de droit. beaucoup a été fait pour accueillir ces élèves différents et les intégrer au mieux au sein des classes. L'instauration, en 2000, d'auxiliaires de vie scolaire, ou AVS, désormais devenus accompagnants des élèves en situation de handicap, ou AESH, a été une étape charnière. aujourd'hui totalement inenvisageable d'imaginer scolariser des enfants handicapés sans l'aide d'AESH ; au contraire, bien des parents, mais aussi bien des enseignants, déplorent le nombre insuffisant de ces professionnels, dont le statut et la formation sont à préciser. La dignité et la grandeur d'une société se mesurent notamment à l'attention accordée aux plus fragiles et aux moins chanceux. Certains ont tendance à toujours voir le verre à moitié vide,

on peut faire mieux, et on doit faire mieux, mais je le dis à ceux qui doutaient de la pertinence et de l'efficacité de l'exercice parlementaire, ce texte, amélioré sur de nombreux points par la commission de la culture du Sénat, est un bon exemple des vertus du bicamérisme. J'espère donc

Laurence Cohen, sur l'article. Permettez-moi de relever un paradoxe, monsieur le ministre. Le gouvernement auquel vous appartenez a engagé, en octobre dernier, une concertation intitulée « Ensemble pour une école inclusive ». Vous parlez de l'école inclusive comme d'une priorité, et nous partageons vraiment cet objectif, mais vous continuez à maintenir dans une forme de paupérisme, sans aucune reconnaissance, le personnel indispensable à la scolarisation des enfants en

la demande de prise en charge, d'accompagnement et de rééducation de ces enfants en situation de handicap. Il convient donc d'avoir une ambition beaucoup plus grande que celle que vous portez au

toutes ses imperfections- si nous en parlons encore aujourd'hui, c'est que tout n'a pas été résolu du premier coup. L'opposition d'alors comprenait parfaitement que c'était un premier pas, et les familles adhéraient à cet élan républicain.

Il serait très regrettable que l'on prétende que ce gouvernement ne souhaite pas la plénitude de l'école inclusive, ne souhaite pas faire le maximum pour les élèves en situation de handicap ; c'est tout le contraire

Ainsi, grâce aux débats d'aujourd'hui, nous pouvons remettre les choses sur les rails, et toute personne de bonne foi souhaitant la réalisation d'une école inclusive meilleure doit adopter cette tonalité, qui permet d'améliorer les choses par le dialogue. La concertation a produit des éléments extrêmement intéressants. D'abord, elle a conduit au constat d'une relative inefficacité de notre système et d'une relative frustration. Beaucoup a été accompli depuis vingt ans, mais ces accomplissements sont insuffisants

Cette transformation est déjà, en soi, un progrès, mais elle n'est pas un progrès suffisant, dans la mesure où, très souvent, les AESH sont à temps partiel et que leur rémunération reste, dans

que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ou CDAPH, dont ils dépendent a validé un accompagnement rendant cette scolarisation possible. Il paraît donc nécessaire d'inscrire dans la loi que les décisions de la CDAPH s'imposent

En effet, les décisions de la CDAPH reposent sur des évaluations effectuées par les équipes pluridisciplinaires des maisons départementales des personnes handicapées,

évaluations sont ensuite validées par la CDAPH, qui comporte des élus départementaux, des représentants de l'État, notamment de l'Éducation nationale, des organisations syndicales, des associations, des parents d'élèves, ainsi que des représentants des personnes handicapées et de leur famille. Cet amendement tend donc à prévoir que les équipes de suivi de la scolarisation existant dans chaque département ne se borneront plus à assurer seulement le suivi des décisions de cette commission, mais les feront appliquer à la lettre,

Ma chère collègue, je suis d'accord avec le début de votre intervention : les décisions de la CDAPH s'imposent. C'est la loi.

Il s'agit de prévoir qu'un décret en Conseil d'État précise le volume horaire et le cahier des charges des contenus de la formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants en situation de handicap handicap délivrée aux enseignants et autres personnels de l'éducation nationale, dans le cadre tant de leur formation initiale que de leur formation continue. Il semblerait en effet

de la commission ? Le Gouvernement dispose déjà d'un pouvoir réglementaire autonome en la matière. Par ailleurs, à l'article 12 , nous avons déjà prévu qu'un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique dispensée aux personnels enseignants et d'éducation en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap. Cet amendement lui semblant en grande partie satisfait, la commission émet un avis défavorable. Quel est

Il peut ainsi apparaître inadéquat de développer l'école inclusive sans comptabiliser ces élèves dans les effectifs de leur classe. Alors que la politique de dédoublement des classes se généralise, donc les créations de postes, arguer

récente. À mes yeux, il est évident que les élèves des ULIS doivent être comptabilisés à l'école primaire, au collège et au lycée,

l'amendement n° 132. Cet amendement, comme le précédent, vise à empêcher la généralisation des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, les PIAL, introduite par ce projet de loi alors même que les expérimentations en cours n'ont donné lieu à aucune évaluation.

Outre que cette modalité d'accompagnement est très difficile à appliquer, notamment dans les zones rurales où les établissements sont trop éloignés, les mutualisations se traduisent, là où elles sont déjà mises en oeuvre, par une dégradation très importante de la qualité de l'accompagnement. Dans un contexte austéritaire où l'offre d'accompagnement est bien souvent inférieure aux besoins, les AESH se retrouvent à devoir arbitrer entre les élèves pour savoir à qui ils consacreront leurs heures, par exemple lorsque celles-ci se chevauchent dans les emplois du temps. La mutualisation conduit en fait, le plus souvent, à réduire le temps de suivi et à dégrader la prise en charge. Quant à l'apport d'un tel mécanisme pour les accompagnants, si l'objectif est d'améliorer leur situation, force est de constater que le moyen est contre-productif. Partout où elle est déjà mise en place, la mutualisation mène à une dégradation des conditions de travail : les trajets entre établissements

La mutualisation ne permet ni un meilleur accompagnement ni de meilleures conditions de travail pour les accompagnants. Son objectif est purement comptable : elle permet de rationaliser à l'envi l'accompagnement et de donner à sa gestion une plus de partir des besoins, mais de se partager les moyens alloués dans un contexte de pénurie. Cette logique est aux antipodes de l'ambition de la loi de 2005. Le sujet de l'école inclusive mérite mieux- nous sommes tous d'accord sur ce point. Ne nous satisfaisons pas de simples solutions comptables aux conséquences sur le terrain souvent désastreuses. La

après la discussion en séance d'une proposition de loi socialiste portant sur le même objet. Le dispositif du Gouvernement était donc déjà rédigé au moment de la restitution de la concertation, alors même que certains sujets étaient loin de faire l'unanimité parmi les participants-

gestion rigoriste, trop économique, des AESH, et que l'aide individualisée ne soit réduite au profit d'une généralisation de l'aide mutualisée. Nous avons rencontré des AESH ; ils nous ont indiqué qu'actuellement,

que des instruments de gestion comptable, non des outils en faveur d'une réelle politique de scolarisation.

au sein des écoles, notamment en milieu rural, n'a pas été précisé, alors que les temps de trajet entre plusieurs écoles risquent d'affecter l'accompagnement des élèves en situation de handicap et de renforcer la précarité des AESH.

Nous aurions aimé avoir connaissance des évaluations avant toute généralisation. Puisque, toutefois, la volonté politique de M. le ministre est ferme sur ce sujet, nous sommes amenés à vous proposer certaines améliorations et à soulever L'objet de cet amendement est d'apporter certaines garanties à la mise en oeuvre des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, car la mutualisation et le renforcement de la coordination doivent se faire en protégeant les droits des élèves en situation de handicap tout en encourageant la coopération entre les différents acteurs. L'objectif est de transformer les PIAL, aujourd'hui simples instruments de gestion des ressources humaines, en véritables pôles ressource, dotés de moyens adaptés et organisant la coopération entre tous les acteurs, notamment les professionnels de l'éducation nationale formés à cet effet, le champ médico-social et les D'une part, cet amendement vise à préciser que les PIAL sont créés en nombre adapté dans chaque département. En fonction des caractéristiques du département, le nombre de PIAL requis pour couvrir tout le territoire serait susceptible de varier fortement.

s'agit par ailleurs d'associer les enseignants référents au suivi de la scolarité des élèves handicapés, afin de garantir au mieux la coordination.

Nous avons certes pu regretter- nous l'avons dit -l'inscription précipitée de ces pôles dans le projet de loi, à peine quelques mois après le lancement de l'expérimentation, et par voie d'amendement.

que la création des pôles inclusifs d'accompagnement localisés constituait une évolution positive : elle devrait permettre de donner davantage de souplesse à un système qui en a besoin- n'est plus tenable. Elle a aussi l'avantage d'impliquer l'ensemble des acteurs dans l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Voilà pourquoi,

concerne l'amendement n° 446 rectifié de Mme Laborde, la notion de « nombre adapté » est, de mon point de vue, trop floue pour être intégrée dans la loi.

et plus efficiente des accompagnants. Il n'y a pas de raison d'exclure certains handicaps du champ des PIAL. Les élèves souffrant de déficience mentale ou d'autisme peuvent, tout autant que les autres

Tout un discours a été tenu pour dénigrer d'emblée une perspective qui, je le rappelle, est inspirée des meilleures pratiques internationales en la matière. Nous voulons sortir d'un système uniforme, vertical, qui a

Les PIAL ont évidemment une utilité qui va très au-delà de l'enjeu de la mutualisation. Je ne répète pas ce que j'ai dit, mais je pense notamment- cela a été dit par M. le rapporteur -aux effets de réseau, qui sont extrêmement importants.

et d'autres établissements scolaires de son environnement, mais aussi entre le collège et les instituts médico-sociaux. Je l'ai dit, et ce point est extrêmement important : nous évitons les effets de cloisonnement ou de « bulle » qui ont pu exister jusqu'à présent.

je souscris à une grande partie des propos qu'elle a tenus, qui, d'une certaine façon, illustrent ce que je viens de dire, c'est-à-dire le besoin de disposer de toute une série d'éléments précis

Sur le fond, je crains que cette mesure ne nuise gravement à l'accompagnement des enfants en situation de handicap et n'améliore aucunement la situation des professionnels d'accompagnement. En cela, je partage l'inquiétude des familles et des collectifs d'AESH, ainsi que leur incompréhension. Comme eux, je crains que ces pôles soient généralisés uniquement pour permettre une mutualisation forcée des AESH. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas de s'opposer à l'idée de mutualiser les expertises néanmoins, nous savons d'expérience que nombre d'élèves en situation de handicap sont fragiles, vulnérables, et qu'ils ont besoin, à ce titre, d'une aide individualisée, qui s'inscrive dans la durée. Ces enfants doivent pouvoir être accompagnés par une personne qui leur donne confiance en eux, les sécurise et leur permette de grandir. à notre sens, ouvrent la voie d'une mutualisation des AESH qui ne répond pas aux besoins spécifiques d'un accompagnement individualisé. Les retours d'expérience du terrain tendent à montrer que la mutualisation met en difficulté à la fois les enfants, qui ne bénéficient pas d'une aide suffisante, et les AESH, qui se retrouvent en responsabilité pour déterminer la quotité de temps à effectuer auprès de tel ou tel enfant.

Le scrutin est ouvert.

est ainsi libellé : La parole est à M. le ministre. Conformément à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, est seule compétente pour notifier un accompagnement humain, individuel ou mutualisé. À tout moment de la scolarité de l'élève concerné, la CDAPH peut modifier l'accompagnement initialement notifié, qu'il soit individuel ou mutualisé. En revanche, il n'est pas possible d'effectuer ce changement en moins de quinze jours, car les procédures de demande de modification auprès de la CDAPH ont des délais incompressibles de traitement, pour une démarche de qualité.